Dans la discussion générale, la parole est à M. Jérôme Durain, auteur de la proposition de loi. Monsieur

Cette avocate écossaise s'était fait connaître pour son combat acharné en faveur de la reconnaissance de l'écocide. L'écocide, à savoir la destruction d'un écosystème, est un concept discuté depuis plusieurs dizaines d'années dans le champ juridique international. Quelques pays l'ont intégré dans leur législation nationale, à l'image du Vietnam, particulièrement marqué par la catastrophe de l'agent orange. De Paris à Nairobi, de New York à Sydney en passant par Bangkok, les citoyens du monde entier, en grande majorité des jeunes, se mobilisent pour exiger des gouvernements qu'ils agissent enfin, ou plutôt qu'ils accélèrent leurs efforts, contre le dérèglement climatique. Tandis que les rapports alarmants s'accumulent - un jour sur le climat, l'autre sur l'extinction des espèces -, c'est bien la jeunesse qui se montre la plus responsable en tirant le signal d'alerte. À nous, responsables politiques, d'entendre ce cri d'urgence. À nous d'apporter des réponses concrètes, en nous montrant à la hauteur des attentes des citoyens et des enjeux du XXI siècle. Toutes les solutions ne se situent pas dans le champ législatif, mais c'est bien en votant des lois aux philosophies nouvelles que nous pourrons accompagner la société civile dans ce combat qui nous occupera pour les décennies à venir, à savoir la sauvegarde de la planète. Trop longtemps, nous nous sommes reposés sur l'idée selon laquelle les êtres humains étaient assez intelligents et assez raisonnables pour maîtriser eux-mêmes leurs dérives et préserver la planète. Une telle logique témoigne d'un orgueil démesuré. Elle nous a condamnés à l'inaction en matière environnementale. La proposition de loi du groupe socialiste et républicain entend précisément rompre ce cercle vicieux. Elle vise à poursuivre et à punir les crimes les plus graves, qui portent atteinte de manière irréversible à la « sécurité de la planète », pour reprendre les mots de Mireille Delmas-Marty, en inscrivant dans le droit pénal la reconnaissance du crime d'écocide. La notion d'écocide marque l'interdépendance entre les écosystèmes et les conditions d'existence de l'humanité. Le terme d'écocide s'inscrit dans le prolongement direct de la Charte de l'environnement, qui proclame dans son préambule que « l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel L'article 1 du texte définit l'écocide comme « le fait, en exécution d'une action concertée tendant à la destruction ou dégradation totale ou partielle d'un écosystème, en temps de paix comme en temps de guerre, de porter atteinte de façon grave et durable à l'environnement et aux conditions d'existence d'une population ». Les exemples ne manquent pas pour illustrer les conséquences extraordinairement néfastes que peut avoir l'activité humaine sur la qualité de l'air, de l'atmosphère, des sols, des eaux, des milieux aquatiques, de la faune et de la flore. La criminalité environnementale est en croissance. Quoi de plus normal ? Un kilo de corne de rhinocéros peut valoir plus cher qu'un kilo de cocaïne, et fait courir moins de risques aux personnes impliquées. En ce sens, il me paraît bienvenu de redéfinir l'échelle des valeurs protégées. À quelles valeurs la société attache-t-elle une importance toute particulière ? Placer l'atteinte irréversible à l'environnement parmi les crimes les plus graves aurait valeur d'exemple. Avec cette proposition de loi, le groupe socialiste souhaite poser les jalons d'un droit pénal de l'environnement permettant de lutter rigoureusement contre la criminalité environnementale et de punir sévèrement les auteurs de ces actes. Le Sénat a su, par le passé, être précurseur sur les questions environnementales, notamment en faisant adopter la notion de « préjudice écologique » grâce à une proposition de loi déposée par notre collègue Bruno Retailleau. Il s'agit maintenant d'aller plus loin dans le combat pour la préservation de la planète. Avec l'examen de cette proposition de loi, je vous invite, mes chers collègues, à dépasser les logiques partisanes et à faire preuve de responsabilité collective. N'attendons pas qu'une nouvelle catastrophe écologique survienne pour légiférer Cette proposition de loi ne revendique aucune perfection législative. Rares sont d'ailleurs les initiatives parlementaires à pouvoir s'en prévaloir ! Certains, comme Mme la rapporteure, ont reproché à ce texte un manque de précision. D'autres observateurs, que vous avez reçus, madame la rapporteure, jugent au contraire qu'il corsèterait trop le champ d'application de l'écocide et ne serait pas applicable. J'aurais beau jeu de renvoyer ces deux avis divergents dans leurs cordes pour prétendre à une forme d'équilibre législatif Mais les sénateurs socialistes connaissent la nécessité d'aboutir à des lois largement acceptées pour être efficaces. Aussi, je répondrai aux critiques par une main tendue, tant vers la droite de l'hémicycle que vers Mme la secrétaire d'État. Madame la rapporteure, chers collègues de la majorité sénatoriale, le préjudice écologique cher à M. Retailleau avait exigé plusieurs années de discussion et de navette parlementaire pour aboutir. Certains parmi vous ont pointé les progrès que notre législation peut encore accomplir en matière de protection de l'environnement. Dans notre département, madame Mercier, la population avait été choquée par les faibles peines auxquelles avaient été condamnés les responsables de la pollution de la décharge de Montchanin, dont les origines remontent à 1979. La semaine dernière, le pays entier s'est ému de voir Vinci polluer de manière très significative la Seine dans le cadre d'un chantier du Grand Paris. Que risque Vinci ? 75 000 euros d'amende ! Voilà pourquoi nous devons revoir, dans notre pays, l'échelle des peines pour ce qui concerne la criminalité environnementale. Dans mon esprit, Dans mon esprit, la pollution provoquée par Vinci est grave. Elle ne constitue pas pour autant un écocide, qui a vocation à incarner le pire du pire en matière de criminalité environnementale. J'espère d'ailleurs que la qualification d'écocide sera utilisée le moins souvent possible. Le but, c'est que les peines encourues soient dissuasives.

juriste reconnue en la matière, qui souhaiterait objectiver l'atteinte irréversible à l'environnement en s'appuyant sur le concept de limites planétaires. Mme Cabanes, dont l'engagement et la technicité juridique au service de la reconnaissance du crime d'écocide sont indéniables, s'est exprimée à l'ONU le 22 avril dernier à l'occasion de la journée de la Terre. D'autres considèrent au contraire que le droit français existant est suffisant. C'est sans doute la vision défendue par le Gouvernement et l'administration, mais des intervenants reconnus pour leurs compétences en droit de l'environnement nous ont fait part de leur scepticisme quant à cet état de fait. Même après l'adoption du projet de loi pour la reconquête de Notre groupe a d'ailleurs, en la matière, d'autres propositions à avancer ; en témoignera notamment une proposition de loi que Mme Bonnefoy déposera prochainement. Mes chers collègues, les lacunes de notre arsenal juridique encouragent le jeu mortifère de la destruction de l'environnement. Nous nous abstenons de combler ce vide, alors même que nous avons pleinement connaissance des agissements de criminels ou d'entreprises malveillantes. En prenant l'initiative, nous pouvons ouvrir la voie à d'autres pays et à la conclusion de traités internationaux.

obérerait les intérêts économiques de nos champions nationaux. Elle est aujourd'hui prise en exemple en Suisse, en Allemagne et au niveau européen. Surtout, elle contribue, à son niveau, à améliorer les conditions de travail dans les usines textiles du Bangladesh.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, après avoir organisé, en 2015, la COP21, qui a abouti à la conclusion des accords de Paris, notre pays accueille cette semaine, au siège de l'Unesco, des scientifiques et des diplomates issus de plus de cent trente pays chargés d'évaluer l'état de la biodiversité. Qu'il s'agisse du climat ou de la préservation de nos écosystèmes, le même constat alarmant peut être formulé : les activités humaines entraînent une telle dégradation de notre environnement naturel que c'est non seulement notre bien-être à moyen et à long terme qui est menacé, mais notre survie À ces enjeux globaux s'ajoutent des pollutions plus localisées : nous nous souvenons tous de la marée noire de l', en 1999, qui avait souillé les côtes bretonnes ; nous connaissons le problème du déversement de boues rouges en Méditerranée ; nous avons entendu parler, tout récemment, de rejets de béton dans la Seine par un grand groupe de Face à ces multiples atteintes à l'environnement, la France s'est progressivement dotée d'un arsenal législatif étoffé : dès les années 1970, nous avons adopté des dispositions relatives aux installations classées et avons introduit dans notre législation le principe « éviter-réduire-compenser », qui implique d'éviter, dans toute la mesure du possible, les atteintes à la biodiversité et, à défaut, d'en réduire la portée, afin de compenser les atteintes qui n'ont pu être empêchées. Plus près de nous,

Nous travaillons bien sûr dans le cadre défini par la Charte de l'environnement, qui affirme, dans son article 1, le droit pour chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé. Nos collègues du groupe socialiste et républicain proposent aujourd'hui d'aller plus loin en inscrivant dans notre code pénal un nouveau crime d'écocide, dont la définition s'inspirerait de celle du génocide. proposition de loi, le crime d'écocide serait constitué en cas d'action concertée tendant à la destruction ou à la dégradation totale ou partielle d'un écosystème et ayant pour effet de porter atteinte, de façon grave et durable, à l'environnement et aux conditions d'existence d'une population. Ce crime serait puni d'une peine de vingt ans de réclusion criminelle et d'une amende de 7,5 millions d'euros, éventuellement assorties de peines complémentaires. Le montant de l'amende serait multiplié par cinq lorsque l'infraction est commise par une personne morale. Le texte prévoit également de sanctionner la provocation à l'écocide- il s'agit de punir les instigateurs, et pas seulement les exécutants -ainsi que le fait pour un groupe d'individus de préparer un écocide. En outre, par analogie avec le génocide, le crime d'écocide serait déclaré imprescriptible. La commission des lois comprend les intentions des auteurs de la proposition de loi et elle partage leur volonté de sanctionner fermement les atteintes à l'environnement. S'agissant d'un texte de droit pénal, nous devons néanmoins être attentifs au respect de certaines conditions tenant à la précision et à la clarté de la loi pénale, qui sont des exigences de nature constitutionnelle. Or les travaux que j'ai menés au nom de la commission ont montré que la rédaction de ce texte souffrait de trop d'imprécisions pour que l'on puisse déterminer en toute rigueur à quelles situations il trouverait à s'appliquer. D'une manière générale, le texte n'opère pas de distinction entre activités légales et illégales : il donne l'impression qu'une entreprise dont l'activité dégraderait l'environnement pourrait être poursuivie quand bien même elle se conformerait scrupuleusement à toutes les prescriptions réglementaires en vigueur. Tel qu'il est rédigé, le texte n'indique pas clairement si la dégradation de l'environnement doit être le but recherché par les auteurs de l'infraction ou s'il peut s'agir d'une conséquence de leur activité, ce qui couvrirait un champ beaucoup plus large. La proposition de loi fait en outre référence à des notions qui paraissent bien floues comment apprécier les limites d'un écosystème ? Qu'entend-on par « atteinte grave et durable à l'environnement » ? Que vise la référence aux conditions d'existence d'une population et comment déterminer les contours de cette population ? Outre cette critique interne, il convient de s'interroger sur l'apport de ce texte au regard des dispositions de droit pénal de l'environnement déjà en vigueur. Il ne nous semble pas qu'il existe aujourd'hui de lacune dans notre droit positif qui rende indispensable la création de ce crime d'écocide nos services de contrôle et nos tribunaux disposent de tous les outils juridiques pour sanctionner les atteintes à l'environnement commises sur notre territoire. Le code de l'environnement comporte déjà de nombreuses incriminations pénales qui permettent de sanctionner, par exemple, les rejets polluants en mer, les atteintes au patrimoine naturel ou à la conservation des espèces, la pollution des eaux, le rejet dans l'atmosphère de substances polluantes ou la mauvaise gestion des déchets. Par ailleurs, des incriminations pénales plus générales peuvent être utilisées pour réprimer les atteintes à l'environnement lorsque des individus en sont victimes, par exemple le délit d'atteinte involontaire ayant entraîné la mort ou celui de mise en danger de la vie d'autrui. Je souligne également que les pouvoirs publics ont à leur disposition une palette de sanctions administratives qu'ils peuvent utiliser pour mettre un terme à des infractions environnementales : un exploitant peut être mis en demeure de se conformer à ses obligations, sous peine de sanctions financières, sans qu'il soit nécessaire de saisir le juge pénal. Dans ce contexte, notre commission est arrivée à la conclusion que l'introduction dans notre droit d'une nouvelle incrimination de portée générale, aux contours assez flous, ne s'imposait nullement. Il nous paraît préférable de mobiliser d'autres outils pour renforcer la protection de l'environnement, à l'échelle internationale et dans le cadre national. À l'échelle internationale, la France pourrait par exemple oeuvrer en faveur de la conclusion d'un traité définissant un socle de sanctions, lesquelles seraient ensuite déclinées dans le droit interne de chaque État partie, afin d'encourager ceux dont la législation environnementale est la moins développée à se rapprocher des meilleurs standards. Une telle approche serait cohérente avec les réflexions développées au sujet de l'écocide par certains universitaires, qui appellent de leurs voeux une évolution du droit international. Dans notre pays, nous pouvons certainement renforcer les moyens de contrôle afin que nos règles environnementales soient mieux respectées. Sur ce point, le projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité et de la chasse, adopté par le Sénat le 11 avril dernier, contient des mesures techniques intéressantes, avec notamment le rapprochement de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et le renforcement des pouvoirs des inspecteurs de l'environnement. Je signale également qu'une mission conjointe du ministère de la justice et et du ministère de la transition écologique a été lancée en 2018 pour améliorer l'application du droit de l'environnement, notamment en renforçant la formation des magistrats et en mettant à l'étude une meilleure spécialisation des juridictions dans la protection de l'environnement et de la biodiversité.

développer des technologies vertes, etc. Voilà quelques pistes qui montrent que l'on peut être réservé concernant la reconnaissance d'un crime d'écocide sans être partisan de l'immobilisme en matière environnementale. Au total- vous l'avez compris, mes chers collègues -, la commission des lois vous propose de ne pas adopter cette proposition de loi. Si nous sommes conscients de l'urgence qu'il y a à agir sur le terrain de la protection de l'environnement, nous ne sommes pas certains que la solution auteurs de ce texte soit techniquement aboutie, ni même que l'aggravation de la répression pénale soit l'orientation à privilégier dans ce domaine. Nous nous réjouissons néanmoins de l'opportunité que nous donne l'examen de ce texte de débattre dans l'hémicycle de cet enjeu crucial qu'est la protection de l'environnement. Je suis convaincue que de nos échanges émergeront des propositions qui viendront enrichir la réflexion du Gouvernement au moment où s'annonce une mobilisation nationale pour l'emploi et les transitions. je ferai miens les mots de Marshall McLuhan, inventeur du concept de village planétaire : « Il n'y a pas de passagers sur le vaisseau Terre ; nous sommes tous des membres de l'équipage. » La parole

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Jérôme Durain, pour commencer, merci : merci pour cette proposition de loi qui nous donne l'occasion d'aborder un enjeu essentiel,

Or notre droit fondamental est le droit à la vie. Et celui-ci ne peut être garanti si la perte de cette même vie n'est pas elle-même criminalisée. Le droit à la vie va donc de pair avec le fait d'assumer la responsabilité de ne pas tuer. question de la protection d'une vie qui se pose, mais celle de la protection de notre qualité de vie et de toutes les vies qui s'épanouissent sur Terre et doivent pouvoir continuer à le faire. Ainsi le droit de bénéficier d'un environnement sain va-t-il de pair avec la responsabilité de ne pas détruire ce même environnement, pour soi et pour les autres. En prolongeant le raisonnement, la reconnaissance du crime d'écocide s'impose donc, pour Polly Higgins. Cette reconnaissance pénale acterait notre reconnaissance d'un droit à la vie qui serait un droit de la Terre, protégeant les écosystèmes qu'elle héberge et les services vitaux qu'elle nous rend

Ce point, justement, me semble être le point crucial des échanges que nous aurons aujourd'hui : la reconnaissance de notre responsabilité à l'égard de la Terre. Dans ces conditions, un pays peut-il assumer seul une responsabilité attachée aux droits et aux responsabilités de tant d'autres ? Je crois que non.

La lutte contre la criminalité environnementale est une préoccupation constante du Gouvernement. Vous le savez : nous nous appliquons à la renforcer. Je vais vous donner un exemple, parmi beaucoup d'autres-

Je pense également à la mission confiée, le 16 janvier dernier, par le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire et par la garde des sceaux au CGEDD, le pour renforcer l'effectivité du droit de l'environnement. Cette mission va notamment nous permettre d'évaluer l'intérêt d'une spécialisation des magistrats chargés de la répression des atteintes à l'environnement.

néanmoins d'une palette efficace de sanctions et de dispositifs de contrôle, de nature administrative aussi bien que pénale, ainsi que d'incriminations spécifiques- je pense par exemple au terrorisme écologique, à la pollution maritime, aux atteintes à l'environnement commises en bande organisée. Par ailleurs, comme vous le savez, dès lors que les atteintes à l'environnement ont des conséquences pour les populations, certaines incriminations de droit commun relevant du code pénal sont déjà applicables : homicide, blessures involontaires, mise en danger. Aujourd'hui, au regard notamment des exemples qui figurent dans l'exposé des motifs de cette proposition de loi, il me semble que le caractère transnational des faits qualifiés d'écocide justifierait l'adoption d'un corpus juridique international préalablement à la création d'incriminations nationales. est d'ailleurs l'un des objectifs du pacte mondial pour l'environnement que défend le Gouvernement au sein de l'ONU, en mobilisant des États du monde entier.

plutôt imprécise, s'agissant de surcroît d'une qualification criminelle. Qu'entend-on par « destruction partielle » ? Quel périmètre donner à un écosystème ?

du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la justice, qui vise à renforcer le dispositif pénal en matière de criminalité environnementale. Qu'il s'agisse d'un renforcement des incriminations existantes ou d'une réflexion sur la notion d'écocide au niveau international, nous serons attentifs et actifs,

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues, comme vous, madame la secrétaire

« destruction totale d'un milieu naturel ».

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons ce soir tend à insérer dans le code pénal trois nouveaux articles afin de réprimer le crime d'écocide, la provocation au crime d'écocide ainsi que la participation à un groupement ou à une entente en vue de préparer un écocide ou une provocation à un écocide.

Le crime d'écocide serait constitué par « le fait, en exécution d'une action concertée tendant à la destruction ou à la dégradation totale ou partielle d'un écosystème, en temps de paix comme en temps de guerre, de porter atteinte de façon grave et durable à l'environnement et aux conditions d'existence d'une population Ce crime serait puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende. Des peines complémentaires pourraient également être prononcées par la cour d'assises. Les mêmes peines seraient prévues pour les deux autres incriminations pénales, sauf dans l'hypothèse où la provocation à l'écocide n'aurait pas été suivie d'effet, le quantum de la peine se trouvant alors réduit. Pourraient être poursuivies des personnes physiques ou des personnes morales, de grandes entreprises par exemple ; dans cette dernière hypothèse, une peine d'amende, éventuellement assortie de peines complémentaires, serait encourue. Conformément aux articles 113-2 et suivants du code pénal, ces peines pourraient être prononcées en cas d'infraction commise sur le territoire de la République, mais aussi en cas d'infraction commise par des ressortissants français en dehors du territoire. En outre, par analogie avec le génocide, le crime d'écocide serait imprescriptible. On peut s'interroger sur la nécessité d'introduire dans notre législation une nouvelle incrimination, de portée générale, alors que la France dispose déjà d'un arsenal très complet. Les sanctions administratives et pénales existantes permettent aux pouvoirs publics de réprimer l'ensemble des atteintes à l'environnement qui méritent d'être condamnées. Je partage les conclusions de la rapporteure, notre collègue Marie Mercier, car nous disposons déjà de tout l'arsenal juridique nécessaire pour sanctionner efficacement les atteintes à l'environnement. d'État et d'autres orateurs, de négocier une convention internationale définissant un socle de sanctions, lesquelles seraient ensuite déclinées dans le droit national de chaque État partie, afin d'encourager

La sensibilité environnementale est aujourd'hui très prégnante, par le biais de l'école notamment. De nombreuses actions sont menées et le fait de mettre en oeuvre de hauts standards en matière d'écologie peut constituer un facteur d'attractivité pour nos régions.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues, ces dernières années, nous avons pu observer une véritable évolution dans la prise de conscience écologique, à l'échelon tant national qu'international. En septembre dernier, ce sont des centaines de milliers de Français qui manifestaient pour lutter contre le changement climatique. Le 8 octobre 2018, nous prenions connaissance du dernier rapport du GIEC, qui nous plaçait face à un diagnostic effrayant : notre planète connaît une hausse des températures de 1 degré depuis l'ère préindustrielle, et le réchauffement climatique progresse désormais de 0,2 degré par décennie. À ce rythme, la hausse de 1,5 degré pourrait être atteinte entre 2030 et 2052, avec des conséquences dramatiques pour les systèmes naturels et humains dérèglements climatiques et multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes ; fonte des glaces et, en conséquence, montée du niveau de la mer ; raréfaction des denrées alimentaires et de l'eau potable ; risques pour la santé ; développement de la pauvreté ; disparition d'écosystèmes entiers. manière, nous sommes, en outre-mer, à l'avant-garde : nous constatons ces phénomènes en premier. Cette prise de conscience de l'urgence climatique et environnementale face à laquelle nous nous trouvons est également la conséquence directe des scandales environnementaux qui ont fait l'actualité planétaire. Les auteurs de cette proposition de loi, auxquels je tiens auxquels je tiens à rendre hommage, nous révèlent que la criminalité environnementale a tellement augmenté qu'elle est désormais classée au quatrième rang mondial des commerces illicites, après les stupéfiants, la contrefaçon et le trafic des êtres humains. Face à cette hausse des infractions d'atteinte à l'environnement, le présent texte propose la création d'une nouvelle incrimination pénale : le crime d'écocide. Constituerait un écocide « le fait, en exécution d'une action concertée tendant à la destruction ou dégradation totale ou partielle d'un écosystème, en temps de paix comme en temps de guerre, de porter atteinte de façon grave et durable à l'environnement et aux conditions d'existence d'une population ». Imprescriptible, ce crime serait puni de vingt ans de réclusion et de 7,5 millions d'euros d'amende. La provocation au crime, ainsi que la participation à un groupement ou à une entente en vue de préparer un écocide ou sa provocation, seraient punies des mêmes peines, sauf si la provocation n'était pas suivie d'effet. Dans ce dernier cas, le quantum de peine serait plus faible : sept ans de prison et 100 000 euros d'amende.

Or l'impératif de clarté de la loi pénale est une exigence de valeur constitutionnelle, particulièrement lorsque la peine encourue est si élevée. D'après ce texte, le crime d'écocide serait constitué dès lors qu'une action concertée « tendrait » à la destruction ou à la dégradation totale ou partielle d'un écosystème. S'agit-il d'une action qui a pour objectif de détruire un écosystème ou, au contraire, d'une action dont la conséquence en serait la destruction ? À ce titre, le caractère intentionnel est déterminant. De la même manière, la notion d'écosystème n'est pas suffisamment définie. Peut-être aurait-il fallu renvoyer à des notions existant dans le code de l'environnement. Il est également fait référence aux conséquences de cette infraction, à savoir l'atteinte grave et durable à l'environnement et aux conditions d'existence d'une population. le caractère durable de cette atteinte s'entend-il par son irréversibilité ? De même, que vise-t-on par l'expression « conditions d'existence d'une population » ? S'agit-il de l'atteinte à la vie ou à l'intégrité de personnes, ou bien d'un risque ? Enfin, combien de personnes doivent-elles être atteintes pour que l'infraction soit constituée ? Vous le voyez, un grand nombre d'interrogations essentielles se posent.

renvoient à des faits commis à l'étranger. Or- vous le savez -, en matière criminelle, pour que notre pays puisse se saisir de telles infractions, il faut que l'auteur ou la victime soit un Français ou qu'une convention internationale existe. Il arrive également qu'un dommage environnemental affecte plusieurs pays. Dans ce cas, quelle serait la juridiction compétente ? Pour toutes ces raisons, il nous paraît indispensable qu'une réglementation internationale voie le jour, d'autant que notre arsenal législatif, tant pénal et administratif que civil, permet déjà de répondre à l'ensemble des situations rencontrées. S'il ressort des discussions que les poursuites en matière de crimes environnementaux sont rares et que les sanctions sont légères, nous pourrions, comme le propose Mme la rapporteure, encourager les juridictions pénales à se saisir de cet enjeu, pour réfléchir à alourdir certaines peines de façon à les rendre plus dissuasives. La dernière loi de réforme de la justice, défendue par Mme la garde des sceaux, ouvre justement la possibilité de spécialiser certains tribunaux sur des contentieux techniques. Pour conclure, les élus du groupe La République En Marche approuvent évidemment les intentions sur lesquelles se fonde cette proposition de loi et la volonté de lutter efficacement contre la criminalité environnementale. L'inscription de ce texte à l'ordre du jour de notre assemblée a le mérite de prendre acte de la mobilisation de la société et de l'urgence à engager des discussions à l'échelle mondiale.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la rapporteure, mes chers collègues, le 14 mars 2019, les associations Greenpeace, Notre Affaire à Tous, la fondation Hulot et Oxfam attaquaient l'État français en justice afin que celui-ci respecte ses engagements climatiques. Cette action devant les tribunaux, intitulée « l'affaire du siècle », avait été précédée d'une pétition lancée le 17 décembre 2018 et signée par plus de 2 millions de nos concitoyens et concitoyennes. La demande des citoyens et citoyennes se fait forte, et à raison. Les trafics d'espèces protégées ont fait de l'aéroport de Roissy une plaque tournante de la criminalité environnementale. L'utilisation abusive de produits phytosanitaires en faveur d'une agriculture productiviste détruit nos sols et provoque des maladies graves en milieu rural.

Se rendre coupable d'un écocrime revient à attaquer la planète, notre foyer à tous. Mon propre parti, Europe Écologie Les Verts, EELV, appelle depuis plusieurs années de ses voeux un tel ajout dans notre législation. Nous ne pouvons donc que nous féliciter de l'initiative de notre collègue Jérôme Durain et du groupe socialiste et républicain, qui vient combler les lacunes du droit pénal environnemental français. il n'existe tout simplement pas d'échelle des peines en la matière. Certes, des contraventions sont prévues pour répondre aux incivilités que commettent certains particuliers, en jetant des détritus ou en braconnant, de même qu'il existe des sanctions administratives à l'encontre de certaines entreprises coupables de délits polluants. Toutefois, parmi elles, le nombre de sociétés mises en demeure reste résiduel. Pour l'heure, il n'existe pas de réponse pénale adaptée à la criminalité industrielle des grandes entreprises, qui bénéficient de l'adage. Pour les

Néanmoins, même si cette proposition de loi était adoptée, que pourrions-nous faire à l'échelle nationale si un nouveau Fukushima se produisait ? Que pourrions-nous faire contre le braconnage de masse des rhinocéros en Afrique, tués pour leurs cornes ? Comment pourrait-on sanctionner Bolsonaro, qui prévoit de bétonner l'Amazonie, poumon vert de la Terre ? Rien de bien concret. Pour sauver l'environnement, la réponse devrait être transnationale et supranationale. L'écocide mériterait d'être traité au sein d'une d'une chambre spécifique de la Cour pénale internationale, la CPI, comme ce fut envisagé, malheureusement sans succès, lors de la rédaction du statut de Rome en 1998, et comme le préconise d'ailleurs la rapporteure de la CPI dans un document de politique générale datant de 2016. Cependant, compte tenu des obstacles politiques et de la difficile procédure de révision du statut de Rome, il est essentiel que les États incorporent le crime d'écocide dans leur arsenal juridique interne, interne, afin de frayer la voie à une reconnaissance supranationale de cette criminalité. Le Vietnam, qui a depuis longtemps adopté une législation en matière d'écocrime, a ainsi pu interdire, le mercredi 10 avril dernier, l'importation du glyphosate sur son sol. À l'instar des « tribunaux verts » en Inde et de diverses institutions spécifiques qui existent en Nouvelle-Zélande et au Chili, la France aurait tout à gagner à se doter de juridictions et d'un parquet spécialisés dans dans la lutte contre la criminalité environnementale. Selon le dernier rapport du GIEC, nous n'avons plus que douze ans pour inverser la tendance, avant que les dégâts infligés à notre planète ne soient irréversibles. Les multinationales continuent d'agir en toute impunité : depuis 1999, l'entreprise Monsanto est au fait du caractère dangereux du glyphosate, mais elle n'a pas pour autant freiné ses activités. Si nous ne responsabilisons pas ces géants économiques, les générations futures en paieront le prix. Le groupe CRCE soutiendra donc évidemment ce texte. Nous espérons que la droite sénatoriale en fera de même.

cette phrase en anglais, et pour cause, elle a été prononcée hier au parlement britannique, qui devient le premier au monde à voter l'objectif d'urgence écologique et climatique, sur proposition des travaillistes.

ces critiques sont une vue de l'esprit : notre texte vise spécifiquement les actes les plus graves, et les critères pour désigner un écocide y sont clairement délimités. Il s'agit d'une action concertée, qui tend à la destruction ou à la dégradation d'un écosystème et qui porte atteinte de façon grave et durable à l'environnement et aux conditions d'existence d'une population. D'autres, au contraire, nous ont reproché de présenter un texte trop spécifique au vu de ces critères. comme l'a rappelé mon collègue Jérôme Durain, il s'agit de réunir au-delà des clivages politiques pour punir et dissuader les auteurs des atteintes les plus graves à l'environnement. Les entreprises ne sont d'ailleurs pas défavorables à une clarification de notre législation pour

Certes, de nombreuses sanctions existent face à une multitude de possibilités d'atteintes à l'environnement et aux écosystèmes. Mais elles s'inscrivent dans une tradition de sanctions administratives, et ces dernières ne sont plus adaptées aux enjeux actuels ni à l'urgence qui se dessine de plus en plus clairement. Les mafias qui se constituent à l'échelle mondiale et qui font de la criminalité environnementale leur constituent un phénomène nouveau,

-n'est devenu véritablement contraignant et efficace face aux marées noires que lorsque nous avons relevé le quantum des peines après le drame écologique de l'en 1999. C'est alors que l'on a décidé d'imposer des doubles coques aux pétroliers. Ne soyons pas, une fois encore, à la remorque des événements.

En matière de protection de l'environnement et du climat, soyons courageux, comme la France a pu l'être en matière de consécration des droits de l'homme ! Soyons les Lumières de cette lutte contre la criminalité environnementale, ouvrons la voie à des changements aux niveaux européen et international.

Plusieurs têtes de liste aux élections européennes, dont celle de la majorité gouvernementale, se prononcent en faveur de la taxation des transports aériens, dans la continuité de l'audacieuse législation suédoise, qui a évolué récemment. Or l'on nous disait que la convention de Chicago, signée en 1944, ne nous permettait pas de le faire

afin d'étendre la responsabilité des entreprises donneuses d'ordre. Aujourd'hui, elle est reprise par un grand nombre de pays.

tout d'abord dans le projet de loi Égalim, il y a exactement un an, puis dans le dernier projet de loi de finances. Nous attendons toujours la traduction législative de ce dispositif.

ici et maintenant, toute notre responsabilité, à notre échelle, pour reconnaître le crime d'écocide. Madame la rapporteure, à juste titre, vous avez cité McLuhan : « Il n'y a pas de passagers sur le vaisseau Terre nous sommes tous des membres de l'équipage. » Dès lors, avançons ensemble en ce sens : c'est tout notre honneur d'être un pays fer de lance dans la lutte contre les atteintes infligées à l'environnement. Reconnaître le crime d'écocide, c'est se battre contre un possible écosuicide. Avec « l'affaire du siècle », alors que des jeunes se mobilisent et marchent partout dans le monde pour le climat, la question environnementale est au coeur des débats.

chers collègues, que voulons-nous pour notre avenir et celui de nos enfants ? Il faut vraiment conclure. Nous ne pouvons nous permettre d'attendre. Ayons le courage de nous engager sur cette question qui dépasse les clivages politiques : c'est notre responsabilité collective. Jacques Chirac

Les preuves sont incontestables. Notre destruction de la biodiversité et des services écosystémiques a atteint des niveaux qui menacent notre bien-être au moins autant que les changements climatiques induits par l'homme.

Avec la généralisation de la conscience écologique au sein de la société française, de nombreuses voix s'élèvent aujourd'hui pour sanctionner plus sévèrement les écocides, atteintes graves à l'environnement. Ces aspirations rejoignent d'ailleurs d'autres

américain. Il est des risques qu'il faut savoir prendre lorsque l'urgence à agir nous y pousse. La nécessité de protéger notre environnement s'instille durablement dans les consciences françaises, notamment celles des plus jeunes générations, depuis que les premières alertes ont été lancées. L'adoption de la Charte de l'environnement de 2005 a été une avancée supralégislative majeure, qui attend des ramifications législatives concrètes, comme celles que propose le texte examiné aujourd'hui. La doctrine a montré comment, faute d'avancées législatives, nos magistrats fait évoluer progressivement la jurisprudence relative à la notion de préjudice pour permettre l'indemnisation des préjudices écologiques. Nous avons entendu les critiques du texte de Jérôme Durain et de ses collègues, mais il nous paraît quelque peu contradictoire de faire le constat de l'urgence à agir, en citant les rapports du GIEC, qui sont terrifiants, et de considérer, dans le même temps, que les normes en vigueur sont suffisantes et que tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes par le simple renforcement de la formation de nos magistrats ou par l'effet de sanctions, dont on sait aujourd'hui qu'elles ne sont pas assez dissuasives. Ce texte mérite que nous réfléchissions à des améliorations de rédaction plutôt que de le rejeter en bloc. Sur le fond, nous souscrivons aux préconisations des directives européennes qui suggèrent que les sanctions pénales

Nous sommes de plus en plus nombreux à considérer que l'état de dégradation de la planète est tel qu'il est aujourd'hui nécessaire de passer à la vitesse supérieure et de sanctionner pénalement toutes les atteintes à l'environnement, quelles qu'elles soient. Très bien ! Il s'agit de repenser totalement l'agencement de notre droit pénal afin d'y intégrer l'environnement en tant que personne propre. La reconnaissance de l'écocide La reconnaissance de l'écocide revêt plusieurs dimensions juridiques, comme nos amendements tendent à le montrer : elle exige, d'une part, l'élargissement de la notion de génocide afin que des actes de guerre reposant sur des atteintes très graves à l'environnement, comme le recours à l'agent orange au Vietnam, puissent être reconnus comme tels et sanctionnés par la juridiction internationale compétente ; elle requiert, d'autre part, le le renforcement des peines, mais également des moyens et des périmètres d'action de nos juges nationaux, en cas d'atteintes à l'environnement sur notre sol et au-delà, lorsque ces atteintes emportent des externalités négatives mondiales susceptibles de concerner la santé et la qualité de vie des de vie des Français. Ce deuxième point pourrait être satisfait par la création d'une incrimination nouvelle, que nous proposons de modifier, ou par l'élargissement de dispositions pénales existantes, comme la mise en danger de la vie d'autrui. Il ouvre cependant d'autres débats, dont celui qui concerne les modalités de calcul des amendes par les magistrats afin d'éviter les condamnations symboliques et la censure de la Cour de cassation. En conclusion, gardons à l'esprit que ce n'est pas l'écologie qui est punitive- j'en ai marre d'entendre cela ! -, mais c'est la société qui doit l'être, quand une majorité en son sein considère qu'un comportement porte atteinte au bien commun, à l'intérêt général, et à celui des générations futures. Comme le grand débat l'a montré, les citoyennes et citoyens français attendent que nous leur apportions des clés pour agir, et l'action devant le juge pénal en est une. Enfin, si l'action dans le droit pénal français nous paraît nécessaire, légitime et efficace, il faut également intervenir au niveau du droit pénal international, comme le propose la juriste en droit international, spécialiste des droits de l'homme, Valérie Cabanes : « Ne faudrait-il pas reconnaître un crime international qui puisse protéger l'habitabilité de la Terre de certaines activités industrielles nuisibles au climat, à la biodiversité, à la qualité des sols, à l'approvisionnement en eau potable, à l'océan, à la santé

pour rebâtir le vivre-ensemble. Quelle meilleure mise en oeuvre du principe de fraternité que l'ambition de travailler à l'amélioration des conditions écologiques d'existence du plus grand nombre ?

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, force est de constater que les efforts mondiaux pour enrayer le réchauffement climatique et protéger l'environnement ne sont pas suffisants, les collègues qui se sont exprimés avant moi l'ont tous évoqué. En ce sens, le texte proposé a le mérite de nous rappeler l'importance de ce sujet. Cependant, la France n'est pas en reste dans les engagements écologiques que les États doivent prendre en urgence pour limiter les changements climatiques. Depuis 2005, la Charte de l'environnement est dans notre corpus constitutionnel et la France a joué un rôle primordial dans les négociations ayant mené à la conclusion des accords de Paris pour le climat en 2015. Plus récemment, le Sénat a adopté, le 11 avril dernier, le projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité, qui renforce les pouvoirs de police et d'investigation des inspecteurs de l'environnement et des agents commissionnés. La Cour pénale internationale ne reconnaît pas encore de crimes contre l'environnement en temps de paix, mais a encouragé les législateurs nationaux à se saisir de cette question. Dans cette perspective, l'initiative engagée par le groupe sénatorial des socialistes est louable et je remercie notre collègue Jérôme Durain pour le travail accompli, mais les contours de cette proposition de loi ne sont pas bien définis et il n'y a qu'un pas à faire pour affirmer que sa finalité

Dans son article 1, l'alinéa 6 propose une définition de l'écocide qui repose sur la réunion de deux éléments : la présence d'une action concertée tendant à la destruction ou à la dégradation totale ou partielle d'un écosystème

Notre loi doit être précise et non équivoque, selon l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Or la notion d'écosystème est très large. Je cite sa définition courante c'est un « ensemble formé par une communauté d'êtres vivants, animaux et végétaux, et par le milieu dans lequel ils vivent. » Quelles sont donc les limites de l'incrimination, puisqu'il suffit d'une dégradation portant atteinte « de façon grave et durable à l'environnement et aux conditions d'existence d'une population » pour être en infraction ? Quelles destructions sont acceptables, quelles sont celles qui seront qualifiées de « graves » ? La question que je pose ici est de savoir sur quelle évaluation nous devrons nous appuyer pour déterminer une atteinte grave et durable à l'environnement. Quelle échelle de valeurs devrons-nous utiliser ? Il faudrait qu'un acte juridique le précise ou que des articles supplémentaires soient ajoutés à cette proposition de loi. Je ne vais pas évoquer l'expression « conditions d'existence fait également référence à aucune disposition juridique, laissant libre cours aux jugements de valeur et à l'interprétation multiforme du juge. Faisons en sorte qu'une incrimination pour destruction de l'environnement soit suffisamment précise et définie pour être efficace. En tant que législateurs, nous devons nous assurer de l'expression claire et sans ambiguïté de la loi. J'en viens donc à mon deuxième point. Cette proposition de loi n'apporte aucun outil juridique véritablement novateur pour la condamnation des infractions à l'environnement. Notre arsenal législatif s'est beaucoup renforcé ces dernières années et permet déjà de réprimer nombre de ces infractions. La loi sur la biodiversité en vigueur depuis août 2016 a introduit dans le code de l'environnement une définition du préjudice écologique. Depuis cette nouvelle disposition, les atteintes à l'environnement peuvent désormais être indemnisées sur le plan civil. Le code de l'environnement comporte également des incriminations pénales pour poursuivre et sanctionner des actions polluantes, comme le déversement de substances en mer, l'atteinte aux espèces, la mauvaise gestion des déchets ou le rejet dans l'atmosphère de substances polluantes. De plus, des incriminations pénales plus larges, qui existent déjà, peuvent être utilisées pour réprimer les atteintes à l'environnement lorsque les individus en sont victimes. J'ajoute que, dans cette proposition de loi, aucune distinction entre les activités légales et illégales n'est établie. Certaines activités détruisent l'environnement, mais restent dans le cadre réglementaire et légal. Pour illustrer mes propos, je ne citerai qu'un exemple : le projet de mine d'or industrielle en Guyane, soutenu par le Président de la République. L'étude d'impact de 2016, menée par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane, a révélé que l'exploitation de ce gisement provoquerait la destruction de sept hectares de forêt amazonienne et d'habitats naturels, ainsi qu'un fort risque de pollution des cours d'eau. Il n'est, certes, pas acceptable qu'une impunité soit accordée à certaines entreprises. La destruction d'espèces végétales ou animales protégées est intolérable et, par-delà celles-ci, nous devons également être vigilants concernant la destruction d'espèces non protégées.

Doit-on sanctionner de la même manière ces deux cas de figure ? Cela ne me semble ni adapté ni opportun. Une dizaine de pays ont adopté le crime d'écocide dans leur législation, comme le Vietnam et la Russie, cela s'explique par leur histoire. À ce jour, À ce jour, aucune condamnation notoire ne peut cependant être relevée. J'ajoute que, si mettre l'écocide sur le même plan que le crime contre l'humanité ou le génocide, le crime de guerre et le crime d'agression peut sembler pertinent,

Placer sans réserve sur le même plan une destruction des espèces et une destruction méthodique de groupes humains reste contestable. Nous n'avons pas besoin d'un texte symbolique dont la mise en oeuvre est impossible. L'enjeu est avant tout international, trop de conditions sont nécessaires et les failles sont nombreuses qui permettent d'échapper à une incrimination efficace. Cette proposition de loi vise surtout à condamner les actions les plus graves, portant atteinte de manière irréversible à l'environnement.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, l'extension des compétences de la Cour pénale internationale au crime d'écocide, tel que la pollution intentionnelle et durable de l'écosystème au Vietnam, par stratégie militaire, afin d'en affaiblir l'ensemble de la population, est une revendication défendue par de nombreux universitaires

aurait tout intérêt à se montrer force d'initiative sur le sujet, en commençant par inscrire dans la définition nationale du génocide le fait d'y procéder par des atteintes graves à l'environnement, comme ce fut le cas au Vietnam. Plusieurs décennies après la guerre, l'agent orange produit encore des effets dévastateurs sur les générations actuelles des territoires touchés, où de nombreux enfants développent des malformations importantes. Notre droit pénal qualifie déjà d'acte terroriste « le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel ». Ce, à condition qu'il se produise « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ». Ce sont les dispositions de l'article 421-2 de notre code pénal. Pour autant, et chacun en conviendra ici, il est peu probable qu'un juge qualifie un jour le gouvernement d'un d'un État, celui de la première puissance mondiale, d'entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. C'est pourquoi nous proposons de préciser la définition du génocide en complétant le critère « d'atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique » par les mots « par tout moyen, dont l'altération de l'environnement naturel de cette population ». Cette précision tend à allonger la dimension temporelle du génocide, dès lors que ce dernier pourrait être regardé comme tel aussi longtemps que l'environnement naturel restera altéré. L'objectif est de dissuader absolument les chefs d'État de recourir à de telles techniques de guerre.

et son environnement naturel. La précision proposée semble pourtant superflue sur le plan juridique : le code pénal ne dressant pas la liste des moyens qui peuvent être utilisés pour détruire une population,

Cet ajout ne respecte toutefois pas le principe constitutionnel de précision de la loi pénale, la notion d'altération de l'environnement naturel étant particulièrement floue, notamment dans la définition de son intensité. S'agit-il d'une altération grave, durable, ou encore, qu'est-ce qu'un environnement naturel ? En outre, cet ajout ne paraît pas nécessaire, puisque le texte exige une atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique sans préciser le Quel que soit ce dernier, l'infraction sera constituée dès lors qu'il s'agira d'une telle atteinte commise en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe déterminé.

symbolique. En matière diplomatique, la symbolique est beaucoup plus importante qu'en matière législative et disposer d'un tel symbole dans notre arsenal pénal nous rendrait plus crédibles encore sur la scène internationale. Je maintiens

tout en respectant la démocratie dans notre hémicycle. Vous serez majoritaires par des voies artificielles, nous le déplorons, mais nous ferons notre travail pour défendre les intérêts de nos concitoyens.

Le scrutin est ouvert.

affaires qui s'y rapportent ne représentent pourtant que 2 % de l'activité des parquets. Compte tenu du faible effet dissuasif des sanctions administratives, d'une part, et des difficultés que rencontre le juge civil à prononcer des dommages et intérêts, d'autre part, il apparaît comme absolument nécessaire de renforcer notre arsenal pénal. Dans l'attente d'une rédaction satisfaisante de la définition de l'écocide, susceptible de s'appliquer à toutes les atteintes graves et irréversibles à l'environnement, l'adaptation de l'article relatif à la mise en danger de la vie d'autrui pourrait constituer une alternative. On pourrait ainsi étendre son champ d'application aux risques non seulement immédiats, mais futurs, ainsi qu'aux cas ayant donné lieu à une maladie permanente, en plus des mutilations ou des infirmités permanentes. Quel

ensuite, sanctionner la mise en danger, lorsqu'elle expose à un risque de mort, de blessure, mais aussi à un risque de maladie. Dans l'objet de son amendement, notre collègue indique qu'il souhaite avant tout ouvrir le débat. Il me semble en effet qu'une réflexion plus approfondie est indispensable avant d'envisager d'élargir le champ d'application de cet article, qui déborde largement la question de la protection de l'environnement. En visant des risques futurs, en faisant référence au risque de maladie, l'adoption de cet amendement pourrait rendre difficile l'établissement du lien de cause à effet entre le comportement répréhensible et les dommages observés. C'est pourquoi la commission souhaite le retrait de cet amendement ; à défaut

Le scrutin est ouvert.

humain, surtout celui de certaines entreprises peu scrupuleuses, peut avoir sur l'environnement, donc sur les générations futures. Le présent amendement vise à proportionner le montant de l'amende aux avantages tirés de la commission de l'infraction en matière de rejets de substances polluantes dans les eaux. L'amende serait calculée en fonction du chiffre d'affaires de la personne morale. Je tiens à attirer votre attention sur les termes utilisés pour la définition de l'incrimination, ceux dont on nous reproche qu'ils ne seraient pas assez précis pour définir l'écocide, ainsi que sur le fait que la faute non intentionnelle est également retenue par le droit en vigueur. Madame la rapporteure, en ce qui concerne le quantum des peines, vous estimez que les sanctions en vigueur sont dissuasives. Je soutiens le contraire, puisqu'on sanctionne plus aisément des pratiques commerciales trompeuses que des atteintes graves à l'environnement. Les simples arnaques,

nombreux sont les juristes qui donnent l'alerte sur l'inefficacité du droit pénal de l'environnement. Si la reconnaissance du préjudice écologique a constitué une grande avancée et si les sanctions semblent élevées, ce dispositif n'a pas été efficace pour certaines grandes entreprises

de tout ce qui aurait pu être réalisé dans le cadre de cette proposition de loi, de ce que le législateur peut proposer pour revoir l'ensemble du code de l'environnement en vue d'adapter les sanctions aux réalités des dommages causés et au caractère lucratif des infractions environnementales.

Si une réflexion pour rendre les peines encourues par les personnes morales en matière d'infractions environnementales plus dissuasives semble intéressante, il paraît nécessaire de réfléchir à l'échelle des peines de manière globale et non en isolant tel ou tel type type d'infractions. Par ailleurs, en matière d'infractions relatives aux rejets polluants des navires, les amendes prévues par le code de l'environnement pour les personnes morales sont d'ores et déjà importantes, puisque leurs montants peuvent atteindre 75 millions d'euros pour les pollutions les plus graves. De plus, ces amendes peuvent être complétées par des dommages et intérêts très substantiels, notamment pour préjudice écologique, ce qui a nécessairement un effet dissuasif pour les entreprises. Pour ces raisons,

et la peine encourue. Ainsi, dans une décision de 2013, le Conseil constitutionnel a censuré la fixation d'un montant maximal de peine encourue dépourvu de lien avec l'infraction à laquelle il s'appliquait, parce qu'il était fondé sur le chiffre d'affaires.

de l'environnement et du développement durable sur la politique pénale en matière environnementale de la France devrait rendre ses conclusions en septembre prochain. Dans ces conditions, monsieur

Le présent amendement, dont nos collègues Josiane Costes et Nathalie Delattre sont à l'origine, vise à réaliser une évolution consensuelle à la suite du constat établi par les auteurs de la proposition de loi sur l'importance croissante de la criminalité environnementale dans les profits des réseaux de délinquance et de criminalité organisées.

de manière directe ou indirecte. Le sujet est d'ailleurs pris très au sérieux par Interpol, qui a adopté plusieurs résolutions depuis les années 1990 pour combattre ce phénomène dans toutes ses dimensions criminalité liée à la pêche, criminalité forestière, criminalité liée à la pollution et aux espèces sauvages. Afin de renforcer nos juridictions dans la lutte contre la criminalité environnementale, il est proposé de permettre à nos magistrats de disposer des moyens d'enquête et d'instruction prévus à l'article 706-73 du code de procédure pénale pour parvenir à sanctionner les délits prévus par le code de l'environnement.

mais à renforcer davantage les moyens à disposition des magistrats dans les cas déjà prévus et à étendre le dispositif à tous les délits du code de l'environnement. Ces évolutions nous paraissent absolument nécessaires pour nous prémunir contre une spécialisation des réseaux de criminalité organisée dans des activités non respectueuses de l'environnement, ce qu'on observe déjà chez certains de nos voisins européens, par exemple en matière de traitement des déchets. Quel est l'avis

organisée. Les enquêteurs et magistrats disposent de pouvoirs renforcés en matière de lutte contre la criminalité et la délinquance organisées. Ils peuvent mettre en oeuvre des techniques particulières de surveillance, d'infiltration, d'enquête sous pseudonyme, d'interception des correspondances et de sonorisation des véhicules, véhicules, potentiellement attentatoires à la vie privée. De plus, des règles dérogatoires s'appliquent en matière de garde à vue comme de perquisition. Il nous paraît hasardeux d'étendre, sans avoir procédé au préalable à une réflexion approfondie, le champ de ces techniques potentiellement très très intrusives à des délits aussi nombreux et d'une gravité variable. J'ajoute que certains délits environnementaux peuvent déjà donner lieu à l'utilisation de ces techniques d'enquête. En effet, l'article 706-73-1 du code de procédure pénale vise notamment les délits d'atteinte au patrimoine naturel

son adoption permettrait l'utilisation de techniques spéciales d'enquête comme les, la sonorisation ou la captation de données informatiques pour les délits prévus par le code de l'environnement, dont certains ne sont sanctionnés que par une peine d'amende.

Il y a une exigence de cohérence. Quant au scrutin public, il ne s'agit pas d'un vote solennel, mais d'un mode de votation qui permet à chacun d'entre nous de prendre ses responsabilités en exprimant son choix sur les amendements.

Comme le prévoit la Charte de l'environnement, « l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ». Il convient donc de doter nos institutions judiciaires des moyens de lutter contre les atteintes à ce patrimoine commun exploitées par des réseaux de délinquance et de criminalité organisées là où elles adviennent,

compétentes pour juger les personnes résidant habituellement sur le territoire de la République qui auraient commis à l'étranger un crime ou un délit en bande organisée accompagné d'une atteinte à l'environnement. Actuellement, des poursuites sont possibles pour des faits commis à l'étranger en cas de crime contre humanité ou de crime de guerre, à condition qu'aucune juridiction nationale ou internationale ne demande l'extradition de la Je comprends bien l'intention des auteurs de cet amendement, qui souhaitent affirmer la détermination de la France à lutter contre les atteintes à l'environnement, même lorsqu'elles sont commises à l'étranger. Néanmoins, je me dois de signaler les difficultés diplomatiques et pratiques qui résulteraient de l'adoption d'une telle disposition : la France pourrait se voir reprocher de s'ériger

D'abord, il ne semble pas conforme aux exigences de précision de la loi pénale. Ensuite, pour que la compétence extraterritoriale française soit effective, il est nécessaire, comme le prévoit l'article 689 du code de procédure pénale, qu'elle soit adossée à une convention internationale reconnaissant les mêmes infractions.

et durables infligées à la faune et à la flore par les activités humaines. Reste que, comme je l'ai souligné dans la discussion générale, pour que de telles sanctions soient efficaces et effectives, elles devront à l'avenir devenir dissuasives à l'échelle supranationale, en s'incorporant dans les statuts de Rome de la Cour pénale internationale, la pour qu'une telle introduction dans le droit pénal international soit possible, il semble nécessaire de trouver une qualification des crimes environnementaux susceptible de convenir à tous les États membres de la CPI. En tant qu'historienne, je me suis interrogée sur la sémantique du terme « écocide ». S'agit-il du bon mot ? Celui-ci est-il adapté et proportionné ? Ne rappelle-t-il pas trop la notion de génocide, ce qui pourrait déplaire à certains États, comme l'Allemagne, ou l'Arménie ? Ne faut-il pas prendre en compte les sensibilités historiques des nations face à un terme si lourd de sens ? Une telle formule ne serait-elle pas considérée comme susceptible de desservir la lutte contre les préjudices environnementaux, en lui donnant le même seuil de gravité que le génocide ?

J'ai pris en compte toutes ces considérations et suis finalement arrivée à la conclusion que l'écocide est entré dans le vocabulaire des associations et des experts. On ne peut pas aller contre le chemin parcouru par les mots, qui, comme des cailloux, roulent à leur rythme et font leur chemin. La

L'homme, par son égoïsme trop peu clairvoyant pour ses propres intérêts, par son penchant à jouir de tout ce qui est à sa disposition, en un mot par son insouciance pour l'avenir et pour ses semblables, semble travailler à l'anéantissement de ses moyens de conservation et à la destruction même de sa propre espèce. « En détruisant partout les grands végétaux qui protégeaient le sol, pour des objets qui satisfont son avidité du moment, il amène rapidement à la stérilité ce sol qu'il habite, donne lieu au tarissement des sources, en écarte les animaux qui y trouvaient leur subsistance et fait que de grandes parties du globe, autrefois très fertiles et très peuplées à tous égards, sont maintenant nues, stériles, inhabitables et désertes.

L'écocide permettrait d'apporter une réponse sans appel, d'abord par la symbolique du mot, un véritable électrochoc, et ensuite, parce que, le crime étant inédit, la qualification doit l'être aussi.

ainsi libellé : La parole est à M. Joël Labbé. La consécration de l'écocide dans notre droit interne constituerait un symbole fort, qui permettrait à notre pays de plaider en faveur de sa reconnaissance au niveau international. Pourquoi la France, si prompte à accueillir la COP21 et à vouloir aboutir à la signature de l'accord de Paris, dont nous pouvons être fiers, ne pourrait-elle pas rejoindre les pays

à l'environnement les plus graves, celles qui sont irréversibles et étendues au regard du quantum élevé des peines. Je rappelle de nouveau que la notion d'atteinte à l'environnement n'est pas mieux définie pour les délits prévus par le code de l'environnement en vigueur. Ainsi, constituerait un écocide le fait de porter délibérément une atteinte étendue, irréversible et grave à l'environnement. L'infraction serait également constituée, lorsque l'auteur des faits ne pouvait pas ignorer qu'il pouvait causer une telle atteinte. Le caractère irréversible du dommage qui ne pourra pas être réparé en nature justifie la forte sanction encourue. Cette rédaction s'inspire en partie de ce que la juriste Valérie Cabanes propose en guise d'amendement au statut de Rome de la Cour pénale internationale ; l'intention de nuire ne doit pas être retenue en raison des devoirs que nous avons vis-à-vis des générations futures. L'infraction serait constituée, que l'atteinte soit délibérée ou non intentionnelle, lorsque l'auteur fait preuve d'une imprévoyance consciente. Pour que ces comportements graves puissent être sanctionnés, il convient d'intégrer la responsabilité pénale de l'auteur, y compris lorsqu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement, à l'instar de ce que le code pénal dispose en matière de génocide. qu'il aurait été nécessaire de réfléchir à la gradation de l'ensemble des sanctions prévues par le code de l'environnement, mais le droit pénal environnemental est, en tout état de cause, très en deçà des conséquences graves que certains comportements ont sur l'environnement. Cela explique la teneur de nos amendements en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales. Mme Esther Benbassa. Une politique environnementale courageuse suppose de tenir compte de la mise en péril des conditions d'existence des populations futures. Certains dommages causés par les crimes environnementaux revêtent un caractère irréversible ou de très longue durée, comme dans le cas du chlordécone, un produit insecticide toxique non biodégradable répandu en Martinique et en Guadeloupe dès les années 1970 et qui continue, encore aujourd'hui, de polluer massivement les eaux et les sols. Ces écocides qui menacent l'équilibre de la planète et la survie de l'humanité auront des conséquences directes sur la santé des générations futures, proches et éloignées. Prévenir plutôt que guérir, voilà la ligne directrice qui s'impose à nous, responsables politiques ! Nous avons des devoirs et des responsabilités vis-à-vis des générations futures. Il semble donc fondamental d'insérer le principe de précaution au au sein du crime d'écocide- ce principe est déjà reconnu et consacré par le code de l'environnement et la Charte de l'environnement de 2005. L'ajout de ce principe permettrait la sanction pénale des auteurs au regard des risques encourus de dommages graves et irréversibles à l'environnement, et ce malgré l'absence de certitude scientifique sur ces risques. Sans modifier l'essence du texte, le présent amendement vise donc à ajouter, dans la définition du crime d'écocide, les populations présentes et futures comme victimes de ces préjudices. Quel

Qu'est-ce qu'une atteinte grave ou étendue à l'environnement ? Par sa généralité, elle risquerait, en outre, d'entrer en concurrence avec certaines incriminations beaucoup plus précises figurant dans le code de l'environnement et qui répriment la pollution des sols, de l'air ou de l'eau. L'amendement soulève une autre difficulté : il prévoit qu'une personne pourrait être poursuivie pour écocide, même lorsqu'elle a accompli un acte autorisé ou prescrit par la loi ou le règlement. Il me paraît difficile de faire peser un risque pénal sur quelqu'un qui se serait simplement conformé à ses obligations légales. Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable. 1 rectifié de notre collègue Esther Benbassa et des autres membres du groupe CRCE, il tend à modifier la définition de l'écocide, en précisant que ce crime serait constitué en cas d'atteinte aux conditions d'existence des populations présentes Son objectif est de mieux prendre en compte le droit des générations futures à vivre dans un environnement sain et préservé. Notre commission partage bien sûr cet objectif de protection des générations futures. Elle n'a cependant pas souhaité inscrire dans le code pénal le crime d'écocide pour les raisons que j'ai exposées lors de la discussion générale, qui tiennent notamment au manque de précision de sa définition. L'amendement proposé ne remédie pas à ce manque de précision et pourrait même rendre l'infraction encore plus difficile à cerner.

qui font disparaître des multitudes d'espèces, qui rendent les seuils de particules dans l'atmosphère intenables ou qui rendent les océans trop acides.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande

serait beaucoup plus vaste, donc nettement plus efficace, puisqu'elle ne se limiterait pas aux atteintes à l'environnement perpétrées par les seules bandes organisées, mais à tous les écocides ici définis. Madame la rapporteure, nos magistrats n'ont pas seulement besoin de formation

Le scrutin est ouvert.

Merci